à prévoir une hausse de 10 millions d'euros des crédits destinés aux lignes aériennes d'aménagement du territoire afin de réduire à due concurrence le montant des subventions payées par les collectivités territoriales sur ces lignes. Nos collègues ont soulevé une véritable question : la compensation des subventions consacrées par les collectivités territoriales aux lignes d'aménagement du territoire tout au long de l'année 2020, malgré la faiblesse, voire l'absence de service rendu par les compagnies aériennes concernées en raison de la crise sanitaire.

inclus, en particulier en matière de suppressions de postes, alors que de nombreuses installations nécessitent des interventions humaines. Il nous faudra donc réfléchir à partir de 2023 à un éventuel arrêt de la baisse de sa subvention.

nationaux de 1 million d'euros. La montée en puissance du parc naturel de forêts qui a été créé l'année dernière est complètement absorbée par les agents qui existaient déjà. Il n'y a donc pas besoin de moyens supplémentaires, en tout cas dans l'immédiat.

Cette taxe sur les nuisances sonores aériennes est en chute libre. Sur la période 2020-2021, la perte de financement pour le dispositif d'aide à l'insonorisation des riverains est estimée à l'équivalent d'une année de recettes.

ne baisse pas. Ensuite, la situation des effectifs est plus nuancée que le constat que vous en faites- vous pourrez la retrouver dans le rapport. Si vous ajoutez aux effectifs autorisés ceux qui relèvent des contrats

Monsieur le président, je vais donc m'exécuter et vous confirmer malheureusement que je ne donnerai un avis favorable sur aucun de ces amendements en discussion commune. J'en suis

l'élargissant aux copropriétés, aux propriétaires bailleurs, en intégrant un forfait pour rénovation globale, un bonus, avec des mesures qui bénéficieront d'un financement additionnel de 2 milliards d'euros pour 2021 et 2022. Nous estimons donc que ces amendements sont satisfaits.

nous invitent à ne pas accentuer ce dispositif et même à réduire les montants de C2E attribuables dans le cadre du coup de pouce pour l'isolation des planchers bas.

le chèque énergie. Évidemment, nous partageons le souci de la lutte contre la précarité énergétique. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'a été versée au mois de mai- et que nous prévoyons de verser dans les prochains jours -une nouvelle aide exceptionnelle de solidarité aux ménages vulnérables. La revalorisation proposée aboutirait à une hausse relative du montant du chèque énergie de 27 euros en moyenne. Sa distribution tardive, puisqu'elle interviendrait en avril 2021, ne me permet pas de donner un avis favorable. L'amendement n°

Le Gouvernement a tout de même mis en place un bonus à l'acquisition de vélos à assistance électrique d'un montant de 200 euros, qui vient en complément d'aides qui peuvent être plus locales. Cet amendement conséquence de réduire les crédits en faveur du bonus automobile et de la prime à la conversion et pourrait, c'est une crainte, faire renoncer à l'élargissement du critère d'éligibilité pour la mise au rebut des véhicules classés Crit'Air 3 ou plus anciens. Il remettrait donc en cause l'éligibilité de 50 % des Français au dispositif en réduisant ses moyens. J'émets également un avis défavorable. Par ailleurs, d'autres solutions de mobilité

Pour ce qui est des conditions de ressources, le plafond de revenu fiscal de référence par part est fixé à 13 489 euros, ce qui correspond aux cinq premiers déciles de revenus, donc à la moitié des ménages français, qui sont d'ores et déjà éligibles au bonus. Un relèvement de ce plafond de ressources aurait une incidence sur les finances publiques, sans forcément être beaucoup plus incitatif. Depuis le 1juin 2020, le montant de l'aide a été augmenté ; il est identique au montant de l'aide attribuée par les collectivités territoriales, dans la limite de 200 euros. C'est déjà très incitatif, je pense donc que nous pouvons nous en tenir là.

En complément, et non des moindres, 1 milliard de déciles verts supplémentaires vont également permettre de financer des aménagements cyclables. La Convention citoyenne pour le climat,

défavorable. J'en arrive à l'inventaire des établissements sensibles lancé en 2010 et qui a permis la réalisation de 1 400 diagnostics de pollution. Au regard des obligations des collectivités en matière de qualité de l'air intérieur, vous savez que le Gouvernement a confié confié aux collectivités le soin de poursuivre ces diagnostics, tout en proposant une assistance et une méthodologie qui est aujourd'hui robuste.

Nous excluons toutefois une reprise de la démarche entièrement financée par l'État. Aujourd'hui, nous disposons du cadre et de la méthodologie d'appui, notamment pour les plus grandes collectivités, qui ont tout à fait les moyens humains et financiers de les mener. Nous souhaitons donc rester dans ce champ de compétence.

-et souvent les plus visités. Les préserver, et préserver leur attractivité demande une gestion absolument irréprochable. Le programme 113 bénéficie d'ores et déjà pour 2021 d'une enveloppe de 3 millions d'euros, dont 1,7 million est est consacré à l'inscription de la gestion des biens inscrits, à la réalisation d'études, à la définition du bien et à la clarification des actions à mener en termes de gestion. Une enveloppe de 1,52 million d'euros financera des démarches partenariales proposées aux collectivités, notamment dans le cadre du réseau des grands sites de France.

ont trait à l'accident industriel majeur de Lubrizol et Normandie Logistique. Celui-ci a fait l'objet d'une réflexion de fond, vous le savez, sur les questions d'inspection des installations classées.

30 postes supplémentaires seront ouverts en 2021, et 20 en 2022. Ils seront créés dans les unités départementales, au plus près du terrain. Il nous a semblé pertinent

et économie circulaire. L'Ademe apporte effectivement un soutien indispensable aux collectivités, dans le respect des objectifs de transition écologique et des règles communautaires. Cela étant, le budget et la trésorerie de l'Ademe sont aujourd'hui, semble-t-il, suffisants. Le plan de relance prévoit par ailleurs 900 millions d'euros complémentaires dans le domaine de l'économie circulaire, au bénéfice pour l'essentiel des collectivités locales et de la décarbonation des entreprises. Cette proposition d'abondement supplémentaire me semble donc largement satisfaite.

dans lequel on trouvera 61 millions d'euros consacrés aux investissements permettant de favoriser le réemploi et les solutions de réduction, notamment de substitution des emballages plastiques, l'Ademe a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Citeo, dans le cadre de sa filière REP (Responsabilité élargie des producteurs), appelle les collectivités territoriales et les porteurs de projets qui souhaitent développer des solutions de réemploi à se faire connaître. Par conséquent, si le Gouvernement voit le soutien au réemploi comme un axe important de progrès, il me semble que cet accompagnement supplémentaire

nous avons déjà accompagné cette mise en oeuvre de 12,3 millions d'euros sur quatre ans au titre du fonds pour la transformation de l'action publique. La réalisation de ce projet doit permettre des gains de productivité et un recentrage de l'établissement sur ses missions prioritaires, afin de participer

de son action, au travers de la deuxième stratégie nationale pour les perturbateurs endocriniens ou encore du quatrième plan national santé-environnement actuellement ouvert à la concertation. à la concertation. Une dotation spécifique de 6 millions d'euros a été versée à l'Agence pour la période 2018-2020, afin qu'elle complète son programme de recherche. Une étude de l'alimentation totale sera financée pour évaluer l'exposition des populations par voie alimentaire. par voie alimentaire. J'ajoute que la contribution au budget de l'ANSES est maintenue pour 2021, tant sur le programme 181, à hauteur de 9 millions d'euros, que sur le programme 190, à hauteur de 1,6 million

qui est dans un processus de transformation alliant une réorganisation interne et une modernisation de ses outils d'analyse. Un fonds de transformation pour l'action publique a a participé à cette transition. Une augmentation des capacités de calcul et une mobilisation de technologies innovantes doivent permettre une amélioration de l'observation et de la prévision des phénomènes Une participation à hauteur de 3 millions d'euros sur 2018-2021 doit financer cette transformation. Les évolutions de son organisation interne ont, quant à elles, été soutenues par le fonds d'accompagnement interministériel des ressources humaines, à hauteur de 2 millions d'euros pour 2019-2022. il s'agit d'une volonté d'évolution dans la transition, mais qui doit, si elle gagne en productivité, accompagner une meilleure maîtrise des dépenses publiques. L'avis sera donc défavorable.

Sur ce suivi de la recherche et l'orientation des travaux, je crois que l'ASN bénéficie déjà des de moyens suffisants. Le Gouvernement formule donc une demande de retrait, sinon un avis défavorable. a pour objet la revitalisation des territoires, à laquelle nous sommes évidemment tous très attachés. Depuis 2020, pour les dépenses d'accompagnement à la reconversion économique, notamment des bassins d'emplois touchés par les fermetures de centrales à charbon ou la centrale nucléaire de Fessenheim, deux dispositifs ont été créés : le fonds d'amorçage, qui complète la mobilisation de crédits de droit commun en appui du projet de territoire de Fessenheim signé en février 2019 ; le fonds charbon, qui accompagne la décision du Gouvernement

Compte tenu du délai de maturation de ces projets, la consommation effective des crédits n'a pas saturé la dotation 2020 et fera l'objet de reports sur 2021.

la poursuite de certains travaux et anciens travaux miniers, notamment du pompage, de l'extraction de gaz de mine, de la surveillance des différents sites, du suivi de mouvements de terrain, des travaux complémentaires de mise en sécurité ou même parfois du rachat de bâtiments menacés par des instabilités de terrain.

an interviennent, d'une part, après la réalisation d'importants travaux directement par Charbonnages de France avant sa disparition et, d'autre part, après un soutien à la reconversion des sites miniers financé par l'État, par exemple sur le fonds d'industrialisation des bassins miniers, ainsi que sur des fonds européens, et ce pendant plusieurs décennies. Je crois ainsi que les territoires concernés font l'objet de toutes les attentions et qu'ils sont déjà très largement suivis par l'État. Il ne me semble donc pas nécessaire de mobiliser de crédits supplémentaires.

Les opérateurs jouent évidemment un rôle absolument clé dans notre action en faveur de l'environnement et de la préservation de la biodiversité. D'ailleurs, vous connaissez mes engagements, que je partage avec plusieurs d'entre vous : l'an passé, en tant que parlementaires, nous avons réussi à défendre

pour ne pas diminuer les schémas d'emplois prévus. Aujourd'hui, dans le plan de relance, l'OFB bénéficiera de renforts ponctuels sous forme de contrats de mission. À mes yeux, les projets que nous déterminons

à la création de contrats de mission. La mise en oeuvre du plan, qui est un enjeu majeur pour les collaborateurs de l'Agence, va induire des taxes à haute valeur ajoutée,

des risques, qui développe un contrat d'objectifs et de performance pour 2021-2025, avec des activités clés et des outils d'anticipation des risques qui sont aujourd'hui absolument nécessaires. L'Ineris verra effectivement ses effectifs diminuer de 13 ETP en 2021, soit une baisse de 2,4 %, pour atteindre un effectif plafond de 485 ETP. Toutefois, en tant qu'établissement public réalisant des opérations sur convention avec des opérateurs privés, l'Ineris est autorisé à recruter hors plafond pour réaliser ses prestations. C'est pourquoi l'avis

Contrairement à la situation actuelle, où l'autorisation parlementaire porte seulement sur le niveau des recettes affectées sans regard sur leur utilisation effective, le montant global des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, mais aussi le détail par nature des dépenses effectuées dans le cadre du fonds seront présentés annuellement au Parlement dans le projet annuel de performance.

au FPRNM étaient plafonnées à 131,5 millions d'euros, le Gouvernement a proposé de porter les moyens du fonds à 205 millions d'euros par an, soit une hausse de 56 %. C'est donc la quasi-totalité du prélèvement sur les contrats d'assurance qui sera dorénavant versée au budget général de l'État l'État et ouverte au budget du ministère de la transition écologique. Nous sommes donc- cela devrait vous rassurer -sur un engagement ferme de report de l'intégralité des crédits qui ne seraient pas consommés et d'exonération de gel des crédits du fonds dans la durée du quinquennat.

présentant l'amendement n° II-498, M. Jacquin a interrogé le Gouvernement sur le décret de 1997 qui impose la suppression des passages à niveau sur les lignes ferroviaires fermées depuis plus de cinq ans avant de pouvoir procéder à leur réouverture. Le ministre délégué chargé des transports, qui a présidé le 19 novembre un comité de pilotage sur les passages à niveau, s'est engagé à prendre un arrêté qui permettra la réouverture de lignes avec passages à niveau, dès lors que le niveau de risque est réduit d'un facteur dix, comme le préconise le guide de réouverture de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. Les mesures préconisées par le rapport de la députée Laurence Gayte permettront d'atteindre cet objectif de sécurité à un coût qui est jugé raisonnable.

Madame la secrétaire d'État, je vous demande simplement une compensation de l'État pour l'aménagement de lignes au cas par cas et de façon équitable, au nom de la solidarité nationale avec les territoires les plus enclavés.

Très bien

L'ART a connu une importante extension de son champ de compétences ces dernières années. Elle régule désormais six secteurs, dont l'un, celui du transport ferroviaire, s'apprête à s'ouvrir à la concurrence,

voix l'amendement n° II-98. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite.

en permettant de procéder comme dans les programmes d'actions de prévention des inondations : définir les travaux éligibles et s'appuyer sur les collectivités locales, qui connaissent bien leurs territoires, les constructions et les habitants, notamment pour réaliser des études de diagnostic. Cet amendement ne crée pas de charges nouvelles. Il permet de redéployer, à budget global inchangé sur le programme de prévention des risques, et dans un objectif de simplification, des aides aux travaux de réduction de la vulnérabilité auparavant prévus par les plans de prévention des risques sismiques aux Antilles. Quel est l'avis de la commission Dans le cadre du plan Séisme Antilles, le fonds prend déjà en charge les études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les HLM.

Cet amendement permet de réaliser des travaux de manière volontaire, comme c'est le cas dans les programmes d'actions de prévention des inondations en métropole. Il s'agit donc d'une nouvelle voie de mobilisation du fonds Barnier,

? Cet amendement vise à traduire une mesure qui a été annoncée par le Président de la République dans les Alpes-Maritimes, après les inondations dramatiques de début octobre.

d'être sommée par le Conseil d'État de s'expliquer sur le respect de ses engagements sur la trajectoire carbone à l'horizon de 2030. Nous demandons alors, comme nous le faisons depuis plusieurs années, la remise d'un rapport au Parlement, à compter de 2021, afin de dresser une évaluation du budget au regard des objectifs de la France en matière d'environnement, de biodiversité et de respect de la trajectoire carbone définie. carbone définie. Ce rapport doit intégrer les conséquences des coupes budgétaires et de réduction des effectifs. En effet, aujourd'hui, l'État n'a plus les outils de son ambition et organise sa propre défaillance, en permettant le recours à la sous-traitance et à une perte d'ingénierie évidente. Entre 2009 et 2018, les effectifs du ministère ont fondu de 27 000 emplois équivalents temps plein

est tout bonnement impressionnant. Malgré cette diminution déjà considérable sur dix ans, la réduction se poursuit à un rythme élevé : le plafond des autorisations d'emploi du ministère de la transition écologique, dans le projet de loi de finances pour 2021, est fixé à 36 241 ETPT,

Mon amendement a pour objet que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les conséquences des réductions des effectifs au sein du ministère. Ce document devra notamment étudier les conséquences de la déperdition de transmission des compétences et des savoir-faire, déperdition qui risque de nuire à la mise en oeuvre de la transition écologique au service de l'intérêt général.

Cet amendement vise à répondre à une demande de WWF France, de CLER-Réseau pour la transition énergétique, de la Fondation pour la nature et l'homme et du Réseau Action Climat. de demander la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement établissant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Alors que les collectivités leur champ de compétences en matière de transition écologique et sociale s'élargir, elles ne disposent pas, en particulier les collectivités rurales, des ressources humaines suffisantes pour mettre en oeuvre pleinement les projets nécessaires en la matière. Cette situation est aggravée par la crise sanitaire, qui va engendrer des pertes de recettes significatives pour les collectivités. Considérant par ailleurs la volonté du Gouvernement de faire de l'action locale et de la transition écologique des piliers de la relance, il est urgent d'augmenter le soutien financier de l'État aux collectivités, pour permettre de financer les postes d'ingénierie et d'animation territoriale nécessaires. Cependant, aucun mécanisme à ce jour ne permet de savoir

Pour répondre à l'urgence climatique, il est avant tout nécessaire de réorienter les investissements vers le développement durable. En effet, selon I4CE, les investissements fossiles défavorables au climat représentent plus de 70 milliards d'euros en France et se concentrent principalement dans le secteur des transports. Il faut agir pour que les « investissements marrons » diminuent au profit des « investissements verts », tant privés que publics. Cet amendement a donc pour objet que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur l'élaboration d'une stratégie nationale d'investissement pour accélérer la transition écologique et solidaire. L'objectif est de recenser les investissements publics et privés à programmer pour combler l'écart entre l'investissement actuel et l'investissement jugé nécessaire

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'ai souhaité m'exprimer en amont

pour lequel les prix ont diminué. Mais si les prix ont diminué, c'est parce que la France a pris du retard et que nous avons bénéficié des investissements qui ont été réalisés dans les pays du Nord de l'Europe.

dans les demandes de financement futures réalisées par les opérateurs de la mobilité, de l'énergie, de la construction ou autre, chaque fois que ceux-ci auront besoin de contracter avec l'État. Cette petite économie d'aujourd'hui entraînera, demain, des surcoûts beaucoup plus importants.

que la situation sera examinée au cas par cas, pour chacun des contrats. Vous ne pouvez pas nier, si vous vous intéressez au fonctionnement de la filière photovoltaïque, que les producteurs historiques, ceux qui ont construit, qui ont installé, qui ont signé le premier contrat avec l'État, sont souvent des sociétés de projet. Une fois que ces sociétés ont pris le risque risque et ont été rémunérées pour cela, elles revendent le contrat à des acteurs qui, eux, détiennent des multitudes de centrales de production. Aujourd'hui, ces acteurs de deuxième rang, qui sont les exploitants,

l'exploitation, j'adresse une simple lettre à mon agriculteur, en lui disant « Cher ami, je ne peux pas poursuivre le contrat », cette simple lettre vaut mutation fiscale. fiscalement titulaire de l'installation photovoltaïque, et l'opération est ainsi faite qu'elle est réalisée pour le prix de revient à neuf. Il existe une déduction de 8 % par an à compter de la dix-huitième année. Les opérations dont nous parlons auront lieu dans ce délai de dix-huit ans. Concrètement, pour un maire que je connais bien dans mon département, la valeur à neuf de l'installation réalisée sur ses grands bâtiments d'élevage représente 4,6 millions d'euros,

qui ne sont pas dotés naturellement de sous-sols riches d'un point de vue agronomique et dont les activités agricoles se déroulent dans des conditions pédoclimatiques très difficiles. Nous venons de vivre une année avec des rendements catastrophiques et des prix qui ne sont pas au

du Gouvernement ? Les 235 000 contrats qui ont été souscrits entre 2006 et 2010 à un prix de rachat très élevé représentent moins de 1 % de la production d'électricité nationale, mais concentrent le tiers le tiers du soutien public aux énergies renouvelables. Afin de protéger les particuliers, les petits agriculteurs et les petites installations, le Gouvernement a ciblé les contrats de plus de 250 kilowatts- ils se reconnaîtront

pèse sur le contribuable, sans déstabiliser l'équilibre financier des installations visées, et pour cause : vous constatez que nous avons introduit une clause de sauvegarde, qui permettra d'observer l'intégralité des impacts économiques sur ces exploitations, de les limiter. C'est une sorte de système de d'alerte. Je le crois, avec ces quelques entreprises qui concentrent le plus gros du soutien public, à des tarifs qui ne sont aujourd'hui plus supportables, nous pouvons nous entendre sur la nécessité de revoir ces relations.

tombent presque ! Et la clause de sauvegarde, je crois que c'est le pompon ! C'est quoi ? C'est la tête du client ? « Toi, tu as droit à l'exonération ; toi, tu n'y as pas droit ! » Il y a un principe d'égalité ; il y a un principe de respect de la parole donnée de l'État ; il y a un principe de réassurance des investisseurs, qui ont qui ont réalisé ces investissements à des moments, comme l'a dit parfaitement Daniel Gremillet, où personne ne savait maîtriser cette technologie. Ils ont donc pris des risques en amortissant un certain nombre d'innovations. Je crois qu'il faut suivre notre rapporteur spécial et l'ensemble de ces amendements pour supprimer vite, au plus vite, cette mauvaise idée.

En outre, il n'y a pas d'appel d'offres. La Commission de régulation de l'énergie, depuis déjà un certain temps, ne soumet pas à appel d'offres. Enfin, on a augmenté la puissance installée sur les toitures, jusqu'à 500 kilowatts-crêtes.

de vote. Je souscris naturellement à l'ensemble des propos de nos collègues sur les risques que fait peser la révision rétroactive des contrats de rachat d'énergie photovoltaïque. De surcroît, alors que le mix énergétique est un enjeu crucial pour l'avenir, la question est particulièrement sensible outre-mer, où le nombre de jours d'ensoleillement fait de l'énergie radiative radiative la principale source de production d'énergie renouvelable, avec un poids significatif dans le mix énergétique. Je ne m'étendrai pas sur le fond, l'essentiel ayant été dit, et je voterai pour la suppression de l'article. Pour autant, je dois le relever, elle ne permettra pas de consolider la clause de prévention des conditions contractuelles du tarif de rachat de l'électricité solaire dans les outre-mer. Aussi, le résultat des travaux de la commission mixte paritaire, je plaide pour qu'ils prennent en compte les conséquences particulières sur les outre-mer, l'idéal étant naturellement que la suppression de l'article soit maintenue.

! Sur le fond, cet article est particulièrement flou. Il évoque la « rémunération raisonnable des capitaux », mais quel est ce niveau ? Y a-t-il un effet de seuil ? Quelles sont les révisions des paliers de rentabilité ? Que dire de la possibilité de recours des producteurs qui pourraient y échapper,

ces crédits. Nous allons procéder au vote des crédits du compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale », figurant à l'état D. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix ces crédits. Nous avons

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous entamons l'examen de la mission « Action extérieure de l'État », dont les crédits s'élèvent à 2,9 milliards d'euros Il s'agit d'une hausse de 66,4 millions d'euros par rapport aux crédits votés en loi de finances initiale pour 2020. Il faut évoquer les importantes ouvertures de crédits survenues en loi de finances rectificative, à

qui ont plus spécifiquement concerné les programmes qu'il traite. Les principaux motifs d'augmentation des crédits en 2021 sont une hausse des dépenses en matière immobilière, pour 27 millions d'euros,

Il s'agira principalement d'opérations lourdes, comme la rénovation des systèmes de climatisation à Riyad ou Djeddah, et de la sécurisation de nos emprises à l'étranger. J'ai été alerté sur le fait que le ministère connaîtrait mal, monsieur le ministre, son parc immobilier, et que la valeur de certains biens n'aurait pas été actualisée depuis l'entrée en vigueur de la LOLF

En ce qui concerne les dépenses de sécurité et les moyens informatiques, elles augmentent de 8,7 millions d'euros, soit 21 % de plus que l'année dernière. La crise sanitaire et le confinement ont révélé des besoins importants en matière de postes informatiques, mais aussi de transmission sécurisée des données. Les dépenses de sécurité augmentent de 7,4 millions d'euros, afin, par exemple, de renforcer le nombre de véhicules blindés ou la sécurité passive des postes. J'en viens aux dépenses de personnel. Malgré les efforts réalisés les années précédentes, le ministère ne respectera pas ses engagements en matière de réduction de la masse salariale et des effectifs. J'estime, à titre personnel, que l'abandon de ces objectifs n'est pas justifiable. Le ministère évoque « une prise de conscience » lors de la crise sanitaire quant au besoin de maintenir les postes. Je constate pourtant que l'un des principaux motifs de non-réalisation de l'objectif cette année est l'augmentation du nombre de conseillers et de personnels supports en cabinet, monsieur le ministre. Au-delà, la masse salariale progresse de 15 millions d'euros sous trois effets principalement : un glissement vieillesse technicité, ou GVT, que nous connaissons bien ici, qui est positif, principalement en raison du recrutement d'agents de droit local, plus expérimentés et donc plus chers une provision pour couvrir le risque prix sur les rémunérations à l'étranger ; une enveloppe de mesures pour la revalorisation des agents de droit local.

de la fin progressive du mécanisme de survocation, qui conduisait à surclasser certains agents de catégorie B et A. À l'inverse, certains sujets n'avancent pas suffisamment à notre goût.

de parvenir à un accord et à une vision commune entre les deux administrations à cet égard. Par ailleurs, contrairement à ce qui constitue ma position personnelle, il n'est toujours pas envisagé d'imposer les IRE

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la suite de Vincent Delahaye, je vais vous présenter les conclusions que je tire, au nom de la commission des finances, de l'analyse des programmes 151 et 185 de la mission « Action extérieure de l'État », qui concernent les Français à l'étranger et les affaires consulaires, d'une part, la diplomatie culturelle et d'influence, d'autre part. Le premier constat, à la lecture du projet du Gouvernement, est la globale stabilisation des crédits alloués à ces programmes, le programme 185 consacré à la diplomatie culturelle augmentant de 2 millions d'euros, soit de 151, consacré, quant à lui, aux Français de l'étranger et aux affaires consulaires, de 0,1 %. Cela traduit, nous l'espérons, la volonté du Gouvernement de maintenir notre influence culturelle dans le monde, notre influence culturelle dans le monde, élément important du rayonnement de la France, et de ne pas diminuer l'attention portée à nos compatriotes dans un moment très sensible, où la pandémie de covid-19 est mondiale. Nous observons, dans cette loi de finances pour 2021, une légère augmentation des moyens du réseau consulaire et de ceux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, Ce budget nous invite toutefois à rester vigilants, tant les acteurs culturels et les opérateurs de notre pays à l'étranger ont été touchés par la crise sanitaire et sociale que nous traversons. Notons aussi que des ouvertures de crédits très importantes ont été décidées cet été, dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 : quelque 50 millions d'euros pour les aides sociales aux Français de l'étranger 50 millions d'euros pour les aides aux établissements scolaires à l'étranger et aux familles non ressortissantes françaises ; 50 millions d'euros pour les bourses en faveur des élèves français à l'étranger ; enfin, 50 millions d'euros d'avances remboursables aux établissements de l'AEFE non portés par la présente Dans ce projet de loi de finances pour 2021, le réseau consulaire évolue très peu, avec un léger recentrage sur la zone indopacifique, pour tenir compte des orientations stratégiques qui avaient été avancées. Le nombre d'ambassades et de représentations permanentes n'a pas diminué depuis 2010, même si le ministère, dans le cadre d'Action publique 2022, dont parlait Vincent Delahaye, s'est engagé dans un plan d'évolution de ses effectifs, un plan d'évolution de ses effectifs, interrompu dans le cadre de ce PLF 2021, tant les postes à l'étranger ont été mis à contribution pour gérer les conséquences de la crise, notamment les rapatriements de très nombreux Français bloqués à l'étranger Les crédits sont, en apparence, stables, mais il faut remarquer que cela masque un double mouvement : une baisse de 2 millions des crédits prévus l'année dernière pour les élections consulaires, sont reportés à 2021, tout comme les élections elles-mêmes ; une augmentation équivalente, soit 2 millions d'euros, des aides sociales en faveur des Français de l'étranger. S'agissant de ces crédits en faveur de l'aide sociale, ouverts à hauteur de 50 millions d'euros dans le PLFR 3, je remarque que seuls 5 millions d'euros ont été jusqu'à présent consommés. Cette consommation très faible témoigne certainement de la difficulté à établir les critères permettant leur attribution, mais nous devrons être attentifs à leur réelle utilisation, dans les mois qui viennent, en fonction des besoins réellement Concernant les moyens consacrés à l'enseignement du français à l'étranger, le Gouvernement affirme qu'il ne renonce pas à son objectif de doublement du nombre d'élèves à l'horizon 2030,

Le budget de l'AEFE s'élève à 1 milliard d'euros, dont 417 millions d'euros dans ce programme, avec une augmentation, notamment, des subventions pour la sécurisation des emprises immobilières. Notons d'ailleurs ici que le recours au compte d'affectation spéciale « Gestion immobilière de l'État » ne s'est pas forcément révélé, l'État lui-même n'étant propriétaire que d'une partie des bâtiments d'enseignement. Ce budget propre est donc bienvenu. En ce qui concerne les bourses, 10 millions d'euros ont déjà été dépensés sur l'enveloppe supplémentaire, et 40 millions d'euros pourraient faire l'objet d'un report, ce qui laisserait une réelle marge de manoeuvre pour répondre aux besoins, en tout cas avec les cas avec les critères actuels d'attribution, à moins que la situation ne s'aggrave profondément au cours de l'année 2021. En ce qui concerne les crédits ouverts en faveur des établissements, la moitié a été consommée, pour l'essentiel au bénéfice des établissements libanais, à la suite de l'explosion qui a touché Beyrouth l'été dernier, plongeant le Liban dans une grave crise. Même si la dotation accordée à Campus France reste, quant à elle, stable, le montant des bourses offertes aux étudiants et chercheurs étrangers diminue de 6 millions d'euros cette année, sous l'effet des restrictions appliquées aux déplacements internationaux. Nous verrons dans les budgets suivants s'il s'agit effectivement d'une orientation contrainte et conjoncturelle liée à la crise sanitaire, qui ne remet pas en cause les objectifs politiques annoncés par le Président de la République et le Gouvernement. L'Institut français voit sa dotation stabilisée, mais il reste confronté à des défis importants, avec le report de grandes manifestations culturelles qui n'ont pas pu se tenir en 2020. Le réseau des instituts à l'étranger, comme celui des alliances françaises,

Enfin, l'attractivité touristique de la France avait, l'an dernier, retrouvé son niveau d'avant les attentats de 2015, mais, dans le contexte de contraction exceptionnelle du tourisme international ces derniers mois, les incertitudes sont encore trop grandes pour lancer de nouvelles campagnes.

Ses crédits devraient encore se réduire davantage pour l'année 2021, à la suite de la chute brutale du nombre de visas octroyés en 2020. En réalité, c'est bien le projet de loi de finances pour 2022 qui sera déterminant pour fixer une nouvelle politique de l'attractivité touristique de la France. France. Disons-le, le budget de ces deux programmes et celui de l'action extérieure de l'État en général sont d'une stabilité qui peut paraître étonnante au regard de l'instabilité du contexte international. Au-delà des reports de crédits de 2020, une nouvelle loi de finances rectificative serait probablement nécessaire si la crise sanitaire et ses conséquences se prolongeaient dans le monde. reconnaissant les efforts faits en 2020, avec un collectif budgétaire très substantiel cet été, je vous inviterai pour ma part et au nom de la commission des finances à adopter les crédits de cette mission. La parole

La pandémie a montré à quel point leur engagement était essentiel ; elle a également pointé les limites des politiques de restriction imposées depuis des années. J'en viens aux défis de sécurisation du réseau français, troisième réseau diplomatique au monde. Outre l'étendue du réseau, la politique étrangère et de défense française, qui se traduit par des interventions extérieures, fait de la France, de ses emprises et des personnels qui y travaillent des cibles privilégiées. La modulation des moyens affectés à chaque poste s'appuie sur le concept de sécurité du réseau

L'avancement du plan quadriennal exceptionnel de sécurisation de 179 millions d'euros pour la période 2017-2020, étendu à 2021 en raison de la pandémie de covid-19, devrait permettre de sécuriser la totalité des emprises dans les pays à risque en 2021.

Le financement par avance du compte d'affectation spéciale 723 est à bout de souffle. Il a permis de répondre à l'urgence, mais présentait trois inconvénients majeurs. il ne finançait que les dépenses relatives à l'immobiliser d'État, ce qui a rendu quasiment impossible l'utilisation des crédits dédiés à l'AEFE. Ensuite, les dépenses éligibles ne concernaient que l'immobilier, empêchant le financement de systèmes de vidéosurveillance pourtant essentiels à la mise en sécurité des emprises. Enfin, et ce n'est pas leur moindre défaut, les avances doivent être remboursées par le versement de 50 % du produit des cessions immobilières entre 2021 et 2025. et 2025. Le retour à 100 % des produits de cession, qui n'est pas inscrit dans la loi, doit être absolument garanti au ministère, et le rythme de remboursement doit être adapté aux possibilités de ventes effectives.

de 207 millions d'euros de votre ministère au désendettement de l'État entre 2014 et 2017. C'est une demande qui a du sens, alors que la vente des bijoux du Quai d'Orsay paupérise l'État.

le champ d'application des travaux de sécurisation des emprises, nous ne devrions pas négliger la sûreté de nos emprises et de nos personnels en Europe et dans le monde occidental en général. Il faut vraiment conclure,

avis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les deux tiers des dépenses du programme 105, que nous examinons ici, servent à financer notre réseau diplomatique et les contributions internationales obligatoires dont s'acquitte notre pays. Dans l'environnement de plus en plus instable que nous traversons, ce sont là des dépenses particulièrement stratégiques. La France n'est pourtant plus qu'au dixième rang des contributeurs des agences de l'ONU, avec une participation annuelle de 1,1 milliard d'euros. Les États-Unis contribuent dix fois plus que nous et le Royaume-Uni, quatre fois plus. Nous sommes même devancés par la Suède, la Norvège et les Pays-Bas ! Parallèlement à l'érosion de notre rang de contributeur, plusieurs États annoncent augmenter leurs contributions, avec l'ambition d'obtenir en contrepartie des postes de responsabilité au sein de ces organisations. La Chine est à présent au sixième rang ; il est d'ores et déjà clair que la France

et des affaires étrangères a saisi l'occasion d'un effet de change positif, qui diminuait de 16 millions d'euros les contributions obligatoires de la France, pour négocier une nouvelle mesure, de 17,2 millions d'euros, au bénéfice de nos contributions volontaires au sein de plusieurs organisations internationales. dépense supplémentaire sera principalement consacrée au renforcement de l'influence de la France dans les organisations dédiées à la sécurité internationale, pour 15 millions d'euros, et à la préparation de l'avenir, pour 22 millions d'euros. Pour la sécurité internationale, des crédits seront dédiés à l'Agence internationale à l'énergie atomique, l'AIEA, dont la France est le sixième contributeur, notamment pour financer des missions de vérification supplémentaires en Iran. Un concours supplémentaire à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, sera consacré en priorité au fonds spécial pour les missions en Syrie, en vue de la destruction du programme chimique syrien. Le fonds de consolidation de la paix de l'ONU bénéficiera quant à lui de 7,5 millions d'euros, au profit d'interventions engagées en fonction des besoins du terrain, notamment dans le Sahel, mais aussi dans les Balkans. Le programme « Jeunes experts associés

d'ores et déjà pour le renforcement et l'inscription dans la durée de cette politique de contribution volontaire supplémentaire, dans le champ du programme 105, car il y a là un signal très positif en faveur du multilatéralisme et de la sécurité. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le retour des politiques de puissance se conjugue avec un affaiblissement du multilatéralisme. Toutes les puissances, grandes et moyennes, ont des stratégies d'influence. La compétition est vive ; une opinion publique internationale émerge. Dans ce contexte, la politique de rayonnement est un volet absolument essentiel de notre action diplomatique. sont dédiés appellent plusieurs remarques. Tout d'abord, la sécurisation du réseau des établissements scolaires et culturels français à l'étranger doit être une priorité absolue.

Nous comptons vivement sur le Gouvernement pour ajuster en gestion ou abonder en cours d'année ces crédits de sécurité, en fonction de l'évaluation des besoins.

En effet, plus de 200 postes ne sont pas pourvus. Est-ce bien le moment de supprimer 71 équivalents temps plein ? La situation est donc critique. Dans ce contexte, le déblocage du système de garantie des prêts aux établissements scolaires est une urgence. Ce système est bloqué depuis plus de deux ans. L'article 48 de ce projet de loi de finances crée un nouveau mécanisme, moins favorable que celui qui avait prévalu jusqu'en 2018 autour l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger, l'Anefe. Le nouveau système plafonne les montants garantis et met fin à la mutualisation des risques entre établissements ; c'est regrettable. Enfin, l'année 2021 sera celle de tous les dangers pour l'ensemble de nos réseaux. La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a ouvert des crédits et avances pour l'AEFE, mais des avances doivent par définition être remboursées, alors que les ressources financières des établissements diminuent. L'enseignement français à l'étranger a en effet perdu 8 000 élèves à périmètre constant. Les instituts français et alliances françaises abordent bien souvent 2021 avec des fonds de roulement à leur étiage, alors que la crise est loin d'être terminée. Nous craignons donc des dommages importants sur nos réseaux l'an prochain, ce qui nécessiterait un nouveau plan de sauvetage semblable à celui qui a été adopté en troisième loi de finances rectificative.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits de la diplomatie culturelle et d'influence appellent de ma part trois observations complémentaires de celles que vient de faire Ronan Le Gleut. En premier lieu, la situation des alliances françaises doit être suivie de très près. Leur enveloppe est strictement identique à celle de l'an dernier, alors que la crise sanitaire les met déjà en grande difficulté. Le réseau compte 832 alliances qui font l'universalité de notre réseau. Hélas, des fermetures sont aujourd'hui probables. En deuxième lieu, les politiques en faveur du tourisme et de la mobilité étudiante devront pouvoir remonter en puissance dès que les circonstances sanitaires le permettront. Une réflexion globale est indispensable : la France a récemment été rétrogradée à la neuvième place pour l'accueil d'étudiants européens. Il faut avoir conscience que nous arrivons aujourd'hui après la Turquie, l'Italie et la Pologne Les bourses jouent un rôle essentiel dans un environnement international de plus en plus concurrentiel. Elles devront remonter rapidement en puissance, et les crédits être intégralement consommés, comme nous le demandons chaque année à l'occasion de la discussion budgétaire.

sur 62 000. Environ 20 millions d'euros d'aides lui ont été attribués, mais il faudra continuer à suivre la situation de très près. Nous souhaitons également que l'aide aux écoles chrétiennes francophones non homologuées soit reconduite. Il s'agit de plus de 300 écoles, qui s'adressent à toutes les catégories sociales sur l'ensemble du territoire libanais.

pour cet exercice budgétaire, nous avons resserré notre focale sur deux sujets. Je traiterai du premier, à savoir la résistance du réseau consulaire et la situation des Français de l'étranger face à la crise sanitaire

et des mesures ont été prises en faveur des 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger, de manière à les accompagner pendant cette période difficile. Des ajustements ont bien sûr été nécessaires, avec le report en 2021 des élections consulaires, du soutien au tissu associatif des Français à l'étranger, le Stafe, et du centre d'accueil administratif mondial, qui est très attendu. Par ailleurs, des crédits additionnels de 100 millions d'euros ont été ouverts en juillet dernier sur le programme 151, dont 50 millions d'euros pour le financement d'un secours occasionnel de solidarité, ou SOS, et 50 millions d'euros pour les bourses scolaires. Représentant 27 % de l'enveloppe initiale, cette majoration est un très bon signal, mais elle ne sera que très faiblement consommée en 2020. Pour 2021, si nous approuvons la hausse de 17 % de la dotation pour l'aide sociale, le principal enjeu dans un contexte sanitaire aussi incertain reste selon nous de disposer des crédits non utilisés de cette rallonge de 100 millions d'euros. Avons-nous été écoutés ? Nous venons d'apprendre que 42 millions des 50 millions d'euros destinés aux bourses seront versés à l'AEFE dès 2020 : tant mieux et merci, monsieur le ministre Pour le secours occasionnel de solidarité, dont le report des crédits est toujours en discussion, il ne faudra pas oublier que cette possibilité a précisément justifié que les crédits du programme 151 n'augmentent pas, contrairement à ceux des autres programmes de la mission. Par ailleurs, la crise sanitaire a renforcé l'intérêt de la dématérialisation de l'administration consulaire. La possibilité de recourir au vote électronique pour les élections consulaires de mai 2021, enfin sécurisée grâce à la reprise de l'entreprise attributaire, qui était devenue insolvable, pourrait se révéler très utile. De même, toutes les dématérialisations de formalités et de procédures offriront certaines économies et facilitations pour les usagers, mais renforceront surtout la résilience des administrations consulaires. Parmi les chantiers toujours en cours en 2021, citons la poursuite de la dématérialisation de l'état civil, la montée en puissance de l'application France Visas et le centre d'accueil administratif mondial joignable à toute heure. Tous les chantiers concourant au consulat numérique doivent être encouragés, mais sans oublier que bénéficier d'un réseau consulaire physique parmi les plus denses au monde- le troisième, pour être exact -s'est révélé un trésor inestimable pour nos compatriotes.

la plus importante des communautés françaises à l'étranger, avec 300 000 personnes, se trouve au Royaume-Uni. À la veille du Brexit, leur situation mérite que l'on s'y attarde. Nous prolongeons ainsi la veille constructive qu'exerce le groupe de suivi de la nouvelle relation eurobritannique du Sénat, initiative commune à notre commission et à celle des affaires européennes. En vertu de l'accord de retrait d'octobre 2019, tout citoyen français arrivé au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 et voulant y rester doit demander un statut de résident- pour une durée de résidence inférieure à cinq ans, au-delà -avant le 30 juin 2021, faute de quoi sa résidence sera illégale. La moitié des Français concernés auraient déjà formulé leur demande, sachant que la procédure, gratuite, dématérialisée et généralement rapide, est ouverte depuis le 30 mars 2019. Hélas, cette procédure entièrement numérisée, impliquant le scannage du passeport et du visage, voire le téléchargement de pièces justificatives, n'est pas accessible à tous. Une demande en format papier reste possible, mais c'est au prix d'un détour procédural plutôt alambiqué. La principale inquiétude concerne les personnes vulnérables, âgées, isolées, ou précaires, ainsi que les enfants placés en famille d'accueil. Heureusement, le consulat de France s'emploie très activement à les identifier. Par ailleurs, les autorités britanniques viennent de garantir que le butoir de juin 2021 sera apprécié avec souplesse et bienveillance. Cependant, une seconde difficulté surgit : la preuve de l'obtention du statut est, elle aussi, dématérialisée, ce qui n'est pas rassurant ; d'ailleurs, notre commission avait déjà déploré cette perspective l'an dernier. Le véritable point d'attention concerne ainsi la période qui suivra le mois de janvier 2021, quand les droits seront différents selon la date d'arrivée au Royaume-Uni- avant ou après le 31 décembre 2020 -, sachant que la preuve de l'obtention du statut ne sera pas exigible avant le 30 juin 2021. Certes, en cas de difficulté, l', instance de suivi de l'application des dispositions relatives aux droits des citoyens européens à partir de 2021, pourra faciliter les échanges avec les représentations diplomatiques et consulaires. Quoi qu'il en soit, nous comptons sur le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, sous couvert de l'Union européenne, pour veiller à ce que la situation des plus fragiles soit préservée, que soit respectée la date du 30 juin 2021 et qu'aucun aléa ne pèse sur les moyens de preuve de la qualité de résident européen.

comme il a déjà été rappelé, l'année 2020 a vu nos réseaux de diplomatie culturelle et d'influence mis à rude épreuve par la crise sanitaire. La quasi-totalité des établissements d'enseignement français à l'étranger, des instituts culturels et des alliances françaises a dû fermer ses portes et réorganiser ses activités à distance. Sur le terrain, les équipes ont fait preuve d'une remarquable capacité de mobilisation et d'adaptation. Qu'elles en soient ici remerciées Les conséquences économiques de la pandémie ont fragilisé un grand nombre de familles scolarisant leurs enfants dans notre réseau d'enseignement et provoqué une forte diminution des ressources propres des établissements.

Nous avons cependant été alertés sur des disparités d'application des mesures, certains postes ayant une lecture personnelle, voire restrictive, des instructions qu'ils reçoivent du ministère. Aussi souhaiterions-nous, monsieur le ministre, recevoir vos explications sur ce qui semble être un problème de communication. Globalement, notre réseau d'enseignement apparaît aujourd'hui en moins mauvaise santé que l'on aurait pu le craindre. La plus grande vigilance s'impose toutefois, d'une part, parce que la situation demeure très instable et évolutive, et, d'autre part, parce que certains établissements sont dans un état plus critique que d'autres. La stabilisation du budget consacré à ce réseau l'année prochaine- hors l'enveloppe spécifique prévue pour la sécurisation des établissements -constitue une garantie importante, mais elle ne permettra sans doute pas de couvrir à la fois les effets de la crise et l'expansion du réseau. Notre commission continue de penser que l'objectif présidentiel de doublement des effectifs est peu réaliste. Surtout, il nous semble que priorité doit être donnée, dans le contexte actuel, à la sauvegarde et à la consolidation des établissements existants. Notre réseau culturel est lui aussi fortement fragilisé. L'incertitude sur les dates de réouverture et sur la capacité des instituts et des alliances à retrouver leurs publics constitue un véritable défi. En l'absence d'amélioration de la situation sanitaire, leurs réserves financières pourraient être entièrement épuisées d'ici au début de l'année prochaine, laissant craindre des fermetures définitives. Le ministère a procédé à des redéploiements de crédits en leur faveur. Cette gestion pragmatique doit être saluée, mais elle ne suffira pas à répondre aux besoins. Monsieur le ministre, envisagez-vous des aides exceptionnelles pour les instituts et les alliances les plus vulnérables ? Sous le bénéfice de ces observations, la commission de la culture a émis un avis favorable à l'adoption des crédits du programme 185. Nous serons toutefois vigilants quant aux conséquences encore non stabilisées de la crise, afin de ne pas laisser des dommages irréversibles atteindre nos réseaux. Mes chers collègues, je vous réseaux. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous le savons, l'exercice comptable est un passage obligé lors de l'examen des missions budgétaires, mais je fais le choix de ne pas m'attarder sur le détail des crédits, que nos collègues rapporteurs ont très bien exposé. Je salue la hausse d'un peu plus de de 2 % des crédits de paiement et des autorisations d'engagement qui sont consacrés à l'action extérieure de la France. J'ose espérer que cette augmentation des moyens de la mission, par ailleurs renforcés au gré des dernières lois de finances rectificatives pour répondre aux conséquences

enfin ! - du schéma d'emploi du quai d'Orsay, après plusieurs années de forte décrue de ses effectifs. Au plus fort de la pandémie, en mars dernier, nous avions mesuré, ô combien, l'importance de conserver des services consulaires efficaces et réactifs, lorsque nos compatriotes installés en dehors de notre territoire sont en difficulté et ont besoin d'être protégés. La sanctuarisation des moyens du réseau diplomatique, le soutien d'urgence à notre diplomatie culturelle, notamment vers l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, ou encore le niveau de nos contributions versées au titre de nos engagements à la sécurité internationale, tout cela, monsieur le ministre, va dans le bon sens Ces choix politiques ont été transformés afin de conforter le rayonnement de la France dans le monde. Mes chers collègues, quittons quelques minutes ces questions budgétaires et permettez-moi de m'interroger sur notre place actuelle dans le monde. Lors de son premier discours de chef d'État, en 1981, François Mitterrand avait déclaré : « Il est dans la nature d'une grande Nation de concevoir de grands desseins. aujourd'hui, les desseins diplomatiques de la France ? À l'occasion de l'examen de la proposition de résolution sur le Haut-Karabagh, j'ai souligné que notre pays a les moyens d'affronter certaines situations, certes complexes, sans se réfugier dans une coupable neutralité. Dois-je rappeler quelques-unes des orientations stratégiques inscrites dans le bleu budgétaire annexé au projet de loi de finances ? On y trouve « Agir en faveur de la paix et de la stabilité », ou encore « Défendre la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit ». Ces axes reposent sur des choix philosophiques qui nous engagent. J'apprécie, monsieur le ministre, les efforts et l'énergie que vous déployez en ce sens. Il vous plaît de rappeler que la France a le devoir de jouer le rôle de puissance d'équilibre. Nous apprécions les difficultés que ce rôle implique dans le contexte géopolitique que nous connaissons, celui du retour des grandes puissances et de son corollaire, la contestation du multilatéralisme. En effet, lorsque la Russie prend la main, si je puis m'exprimer ainsi, afin d'obtenir un cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le groupe de Minsk est marginalisé ; de fait, l'action de la France l'est également. Au Proche-Orient, devons-nous nous contenter d'être transformés en spectateurs passifs, qui assistent, médusés, à la provocante tournée en Cisjordanie occupée de Mike Pompeo, représentant d'un président battu et sur le départ ? En Syrie, la Russie a mis la France hors-jeu. de notre stratégie ? En Libye, le rôle hégémonique, là aussi, de la Russie et de la Turquie nous déclasse. Pis, il nous évince de la séquence diplomatique du règlement d'un conflit aux conséquences migratoires et humanitaires cruelles. En Afrique de l'Ouest, sous peine d'être accusés de renouer avec la Françafrique, nous subissons, impuissants, les aménagements- que dis-je, les arrangements constitutionnels -des présidents sortants désireux de conserver le pouvoir. Enfin, je m'inquiète des timides soutiens de la communauté internationale que la France a reçus face à la colère instrumentalisée d'une partie du monde musulman, plus prompte à dénoncer des caricatures que les persécutions subies par les Ouïghours en Chine.

Dans ces circonstances, il serait temps- nous le répétons déjà depuis trop longtemps ! -que l'Union européenne défende une vraie politique diplomatique : elle est en capacité de hausser le ton, comme elle a su déjà le faire sur les dossiers grec et chypriote face à la Turquie. J'y viens, monsieur le président ! Vous avez souvent déclaré, monsieur le ministre, que l'Europe a les moyens de maîtriser et d'affirmer son destin et qu'elle doit tenir son rôle de puissance d'équilibre. J'ai l'intime conviction que ce moment est arrivé.

Si je ne veux, et ne peux, nier la place de la France dans la diplomatie mondiale, on ne peut être que circonspect lorsque l'on observe l'investissement dévolu à la défense et qu'on le compare à celui de la diplomatie.

rejoint une analyse beaucoup plus récente de l'un de nos ambassadeurs, qui déclarait que « notre diplomatie est en surrégime par rapport aux ambitions du Président. On arrive au bout d'un modèle Ce modèle, on en mesure aujourd'hui le détail, mais aussi les conséquences. En trente ans, le Quai d'Orsay a perdu 53 % de ses effectifs, perte que la précarisation des personnels par le recours à la contractualisation et à l'emploi local n'a pas compensée.

Autre élément positif : les crédits augmentent enfin. On parle, pour cette année, de 66,4 millions d'euros en plus pour la mission, soit une augmentation %. On peut y ajouter les 50 millions d'euros prévus dans le plan de relance pour augmenter la contribution française à différents organismes internationaux, notamment à l'Organisation Malgré cette embellie, notre groupe s'inquiète à plusieurs titres. Premièrement, en dépit de l'activisme, pour ne pas dire des gesticulations, du Président de la République, nous avons le sentiment que la France est de plus en plus inaudible sur la scène internationale. C'est d'autant plus problématique que l'on voit aussi les outils multilatéraux largement affaiblis par leurs divisions internes. Le blocage hongro-polonais du plan de relance européen n'est que la dernière péripétie d'une année 2020, durant laquelle même la crise exceptionnelle du covid-19 n'a pas permis de dégager des horizons communs. Emmanuel Macron et, à travers lui, la France parlent beaucoup. Nous devons lui reconnaître ce volontarisme ! Mais les actes manquent, parce parce que le multilatéralisme est aujourd'hui confronté à des problèmes structurels, mais aussi parce que nos forces diplomatiques ont été affaiblies d'année en année. Deuxièmement, cette timide hausse de moyens ne vient compenser ni les pertes accumulées depuis des décennies ni les besoins exceptionnels de la période. Certes, par à-coups, la France arrive à se démarquer. L'opération de rapatriement de 200 000 de nos compatriotes à l'étranger au printemps a ainsi été remarquable. Quelle réponse pourrons-nous cependant apporter sur le long Je souhaiterais, pour conclure, évoquer le rayonnement culturel de la France. La baisse attendue, mais drastique, de 30 % des étudiants étrangers accueillis en France inquiète.

La France, en suivant les exemples danois et suédois, ne se dote pas d'un outil efficace pour faire face à la concurrence internationale toujours plus forte, et risque le décrochage. Dans la même veine, les 24,6 millions d'euros supplémentaires attribués à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, en accompagnement des 50 millions d'euros prévus par le projet de loi de finances rectificative de l'avance de 50 millions d'euros du Trésor, ne compensent ni la perte de 71 emplois sous plafond ni les surcoûts de la crise, ni la perte des frais d'inscription. À ce titre, je crains que nous ne soyons arrivés au bout d'un modèle du financement par les familles. Au

contre cette mission. La parole est à M. Joël Guerriau. L'année qui s'achève a été particulièrement éprouvante, pour le monde comme pour la France. La pandémie a fortement mobilisé les équipes de l'État au service des Français à l'étranger, qu'ils soient touristes ou résidents. Dès le début de la crise, le ministère a réalisé un travail remarquable qu'il convient de saluer. La crise sanitaire a mis en lumière la nécessité d'accélérer la dématérialisation de l'état civil, en poursuivant le chantier du consulat numérique. En plus de porter une assistance d'ampleur exceptionnelle à nos concitoyens, il a fallu continuer à assurer les missions de diplomatie et d'influence dans un contexte particulièrement dégradé. La pandémie a en effet frappé tous les pays et, ce faisant, a contribué à aggraver les tensions préexistantes sur la scène internationale. Durant cette crise, nous avons vu se poursuivre un recul regrettable du multilatéralisme- tous, ici, vous en avez parlé -, notamment lorsque l'intégrité de l'OMS a été mise en doute par les États-Unis, plus grands contributeurs de son budget. Le président Erdogan, quant à lui, a continué à déstabiliser la Méditerranée orientale et le Levant, mais aussi le Caucase, avivant les tensions partout où il le pouvait. Ces circonstances de crise et de division rendent la diplomatie encore plus nécessaire. Si nous avons de bonnes chances d'en voir la fin au cours de l'année à venir, la situation internationale n'en sera pas pour autant À cet égard, nous soutenons l'augmentation des crédits destinés à l'action extérieure de l'État. La menace terroriste à l'encontre de la France est élevée depuis de nombreuses années et s'est encore renforcée en 2020, comme en témoignent les attaques tragiques de Conflans-Sainte-Honorine, de Nice et Djeddah. Il va de soi que les emprises françaises à l'étranger doivent bénéficier de la meilleure sécurité possible. Ceux qui y travaillent doivent être protégés au mieux, y compris lors de leurs déplacements, lorsque la situation l'exige. À ce titre, nous nous félicitons particulièrement de l'acquisition de véhicules blindés, qui seront plus qu'utiles. Nous soutenons également le renforcement de la sécurité dans les établissements d'enseignement

De même, il convient, comme l'a rappelé mon collègue Le Gleut, de s'inquiéter de l'attractivité de nos établissements d'enseignement supérieur en France, considérant que notre pays occupe désormais la neuvième

Elle s'est encore dégradée avec l'explosion à Beyrouth, qui a détruit une partie de la ville l'été dernier. Nous devons continuer à soutenir ce pays ami dans les épreuves qu'il traverse, sans parler de l'Arménie, dont on a évoqué le cas hier. Nous souhaitons qu'une attention particulière soit portée à ces sujets. L'augmentation des crédits concerne aussi les dépenses de personnel. Le ministère n'atteindra pas les objectifs de réduction de personnel qu'il s'était fixés. C'est certainement dû à l'effort exceptionnel déployé pour la gestion de la crise sanitaire, ainsi qu'à l'enchaînement des crises géopolitiques au cours de cette année, qui bientôt s'achève. Nous notons cependant que l'augmentation de la masse salariale ne peut s'expliquer uniquement par l'inflation, qui lui est très inférieure. Concernant la rémunération des agents, les personnels à l'étranger exercent leurs missions dans des conditions d'éloignement et de sécurité qui justifient parfois le versement d'indemnités, notamment celles de résidence à l'étranger. Notre groupe considère qu'il serait plus juste que le montant de cette indemnité fasse directement partie des rémunérations des agents. Les sommes concernées feraient ainsi l'objet d'une imposition sur le revenu, en plus d'ouvrir des droits en matière d'assurance sociale. Il importe que la rémunération des agents qui travaillent pour la France soit juste et équitable. Cela contribuera à préserver notre réseau diplomatique- le troisième au monde -, qui s'impose comme l'une des grandes forces de notre pays ; il nous permet de promouvoir nos idées, d'entendre celles de l'étranger, et de dialoguer avec tout le monde. est attaché à perpétuer ce modèle. L'année qui s'ouvre s'annonce meilleure que celle qui se termine. De nombreux sujets nécessiteront cependant de mobiliser notre réseau et notre influence. Il est heureux que le temps des réductions budgétaires soit terminé, car il est certain que la capacité diplomatique de la France contribue à sa puissance. Nous devons néanmoins veiller à conserver la force de notre diplomatie. Pour ce faire, nous aurons besoin de continuer à en maîtriser les dépenses, afin de ne pas avoir à abandonner certaines de ses composantes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, la mission « Action extérieure de l'État » présente cette année une stabilité bienvenue. Après avoir perdu la moitié de ses effectifs en trente ans, la diplomatie française connaît enfin un répit. C'est heureux, car, comme le disait un ambassadeur au journal en octobre dernier, « notre diplomatie est en surrégime par rapport aux ambitions du président. On arrive au bout d'un modèle Il faut dire que le Président de la République est partout, que l'activité de la cellule diplomatique de l'Élysée est frénétique et que le Quai d'Orsay a du mal à suivre. La France ne peut pas tout faire, partout dans le monde, surtout avec un budget « à l'os sur les propos précédemment tenus par mes collègues, je précise que les personnels consulaires, comme tant d'autres agents du service public, ont été lourdement sollicités et ont montré à quel point ils étaient indispensables. Il est dommage qu'il faille attendre une crise d'une telle ampleur pour s'en rendre

La suppression de cet objectif de réduction d'emplois constitue une mesure de bon sens, car la crise liée au covid-19 sera toujours d'actualité en 2021. Par ailleurs, je me permets d'appeler l'attention du Sénat sur la question de l'accès aux crédits.

Le bilan de cette ouverture de crédits pose question. Sur les crédits en faveur de l'aide sociale, seuls 5 millions sur les 50 millions d'euros ont été consommés. Sur les 50 millions d'euros ouverts pour les bourses, 10 millions ont été dépensés. Enfin, sur les 50 millions d'euros de crédits ouverts en faveur des établissements, la moitié seulement a été consommée et l'essentiel- il faut le noter -a été mobilisé pour les établissements au Liban à la suite de l'explosion de Beyrouth. Dans le même temps, les effectifs du réseau d'enseignement français à l'étranger ont été amputés de 8 000 élèves environ, à la rentrée 2020.

fragiles. En conséquence, et suite à l'introduction des frais d'inscription différenciés par le gouvernement actuel, le nombre d'étudiants étrangers en mobilité internationale dans les universités françaises baissera de 30 % sur la Il est donc nécessaire d'augmenter les bourses attribuées aux étudiants étrangers afin de rendre l'enseignement français plus attractif. À l'heure actuelle, nos voisins font bien mieux que nous : l'Allemagne, par exemple, prévoit des bourses deux fois plus élevées, tandis que d'autres pays augmentent les montants versés. par l'évocation de la question climatique. Le cinquième objectif de cette mission budgétaire consiste à oeuvrer à une régulation économique et commerciale efficiente, qui soit cohérente avec nos objectifs en matière de développement durable à l'échelle nationale et internationale. Pourtant, ces objectifs, qui représentaient seulement 1 % des crédits

je souhaite réagir à l'amendement n° II-5 déposé par la commission des finances. S'il n'est pas normal que nombre d'ambassadeurs thématiques ne reçoivent aucune lettre de mission, le dispositif des ambassadeurs thématiques ne s'avère pas, en lui-même, problématique. Qu'il s'agisse des migrations, de la Méditerranée, des négociations internationales sur le climat

Ce plan sans précédent joue un rôle d'amortisseur important : aucun autre pays que la France n'a fait preuve d'autant de solidarité à l'égard de ses ressortissants établis à l'étranger, dire. S'agissant des aides sociales, l'accélération du rythme de consommation des crédits ouverts par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 montre que les besoins sont importants et réels ; il faut y voir les conséquences de l'assouplissement des critères d'attribution de ces secours. Quant aux mesures en faveur de l'enseignement français à l'étranger, elles ont permis que la rentrée scolaire se déroule dans des conditions relativement satisfaisantes. Nous pouvons constater une quasi-stabilité des effectifs

découle essentiellement de l'homologation de quatorze nouveaux établissements, qui augure du meilleur pour la poursuite du plan de développement. La crise économique et sociale liée à la pandémie ne fait malheureusement que commencer. Aussi faut-il se féliciter de la prolongation du soutien budgétaire accordé aux Français établis hors du territoire national ; l'augmentation de 22 % des crédits d'aide sociale que je viens de mentionner permettra de faire face.

Je constate avec satisfaction que la priorité donnée à la sécurité se traduit par trois mesures budgétaires, à savoir l'augmentation de 17 % des crédits consacrés à la sécurité à l'étranger, la poursuite de la mise en oeuvre du plan de sécurisation

je note que le projet de loi de finances offre au Quai d'Orsay les moyens d'engager sa révolution numérique. Grâce à l'augmentation de 22 % des crédits consacrés au numérique, les agents du ministère vont enfin pouvoir être dotés d'outils individuels de mobilité- ordinateurs portables, tablettes, etc. ; ils seront ainsi mieux armés

Plusieurs mesures sont attendues par nos concitoyens établis hors de France, à commencer par le déploiement de centres de contact consulaires,

budgétaire ces dernières années. Enfin, je tiens à souligner les bons résultats du Quai d'Orsay en matière de féminisation des postes d'encadrement. En effet, selon un récent rapport

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord, monsieur le ministre, à saluer la qualité de votre engagement personnel, tout comme celui du ministre Jean-Baptiste Lemoyne, à la tête du réseau diplomatique, culturel et consulaire. Les agents de votre ministère méritent aussi toute notre reconnaissance, pour avoir su faire face, avec beaucoup de résilience, tout au long de cette année qui marquera l'histoire.

la concrétisation de l'article 1 de la proposition de loi que j'avais déposée un mois plus tôt, afin que les Français de l'étranger puissent bénéficier de fonds d'urgence mobilisables le fonds d'urgence covid-19. rectificative, vous avez apporté la solidarité nécessaire pour aider les Français de l'étranger se trouvant dans le besoin, en abondant le programme 151 de 100 millions d'euros, avec 50 millions d'euros de bourses supplémentaires et 50 millions d'euros de secours d'urgence. Vous avez également pris en compte la situation des familles en difficulté d'enfants étrangers scolarisés dans notre réseau, lorsque le sénateur Robert del Picchia, le premier, vous a alerté sur cette nécessité. Vous avez ainsi alloué cinquante autres millions d'euros

Depuis lors, ces élus et notre commission ont observé que ce dispositif de solidarité a trouvé un public plus large, grâce à l'assouplissement des conditions d'attribution.

pourriez-vous nous indiquer si la part de ces crédits non consommés en 2020 sur les programmes 151 et 185 sera reconduite en 2021 ? Eu égard au programme 185 portant sur notre réseau culturel et éducatif, chacun reconnaît l'importance de l'AEFE pour la politique d'influence de la France. Depuis vingt ans, cependant, cette influence s'est considérablement réduite. Le différentiel de l'enseignement français par rapport à l'enseignement anglo-saxon à l'étranger était alors de 1 à 3 il est aujourd'hui de 1 à 20. Pour redresser la barre, Emmanuel Macron, d'abord, puis le Gouvernement, par votre intermédiaire, avez fixé l'objectif de doubler les effectifs du réseau d'ici à 2030.

L'audition du directeur de l'AEFE a démontré que les orientations prises pour son développement peinent à s'aligner sur la vision ambitieuse du chef de l'État. Je n'en suis pas surpris : cette administration se trouve en conflit d'intérêts, car il lui est demandé de développer un réseau précisément destiné à faire concurrence à celui qu'elle administre.

de problème va s'étendre au développement de l'immobilier du réseau. En effet, on apprend aujourd'hui que Bercy confiera à l'AEFE l'instruction des demandes de garantie de l'État sur les prêts relatifs à l'immobilier scolaire, traités auparavant par

Ces diplomates souhaitaient célébrer le premier anniversaire de l'adoption de la résolution sur le Venezuela, que j'avais présentée pour le groupe Union Centriste. Ils voulaient ainsi saluer l'action du Sénat, conforté, sur ce sujet, par le soutien sans faille du président Larcher et du président Cambon.

Pourquoi l'Amérique latine semble-t-elle donc absente du radar du ministère, alors que la France est le seul pays européen à être physiquement présent sur ce continent et que tous nos voisins nous y réclament ?

douze, les citoyens américains résidant en Arabie Saoudite en étaient informés par un message sur WhatsApp. La communication officielle de la France est intervenue, quant à elle, à douze heures trente-trois, tandis que l'information tournait déjà en boucle dans les médias Le 2 novembre dernier, j'avais demandé à Jean-Baptiste Lemoyne que le processus de communication de crise soit formalisé et que nos élus fassent l'objet d'une information spécifique. En effet, lorsque le ministère délivre une information anxiogène, c'est vers ces derniers que nos compatriotes se tournent pour en savoir plus. Pouvez-vous prendre en compte mes inquiétudes sur la pertinence et l'efficacité de notre système d'alerte ? Je tiens à finir par une note positive, monsieur le ministre. Nous sommes à trente-cinq jours de la date fatidique du 31 décembre 2020, qui marquera la fin de la période de transition du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne,

nous refusions de voter un budget qui ne fût pas à la hauteur de nos ambitions, et nous ne voulions pas donner raison à Bercy, qui demande chaque année de nouvelles économies.

je tiens à saluer l'effort budgétaire particulier, qui s'inscrit dans la lignée des gouvernements du quinquennat de François Hollande, pendant lequel la sécurité passive de nos entreprises est devenue prioritaire, puisque 204 millions d'euros lui ont été affectés depuis 2015 un réel effort avait déjà été consenti dès 2013 pour le centre de crise. Je tiens tout particulièrement à saluer le rôle des membres des comités de sécurité et de nos élus locaux, qui se réunissent pour répondre au mieux aux situations locales. Nous pensons néanmoins que des progrès peuvent encore être réalisés en matière de réactivité et de communication en cas d'attaque. Les crédits du programme 151 sont stables. La légère hausse que l'on peut observer est due au report de crédits non utilisés en 2020.

ne relâchons pas nos efforts pour soutenir notre réseau d'écoles francophones et nos établissements de la MLF au Liban. Nous saluons également l'ouverture, pour la première fois, de l'aide aux familles étrangères, qui constituent les deux tiers des effectifs, avec un bémol : celui de la sous-consommation des crédits et de leur non-reconduction en 2021.

Tout comme pour les critères d'obtention des bourses, il me semble urgent de reconsidérer les documents et les informations à exiger des demandeurs ; beaucoup d'entre eux ont fait appel à leurs économies, mais ils risquent de se tourner de plus en plus vers le secours occasionnel.

doit demeurer exceptionnel, d'autant que l'allocation de cet argent public échappe totalement au contrôle des conseils consulaires. Je souhaite aborder maintenant la question des élections consulaires, reprogrammées en mai 2021. Pour désigner les 443 futurs conseillers des Français de l'étranger, près de 1, million de nos compatriotes seront appelés à voter, en présence ou par voie électronique. Or il semblerait que, pour des raisons de sous-effectifs, mais également d'économies, il ait été demandé aux postes de réduire le nombre de bureaux de vote. Si le vote physique est déjà compliqué par la situation sanitaire, comment s'assurer que ces élections se dérouleront dans des conditions satisfaisantes, si, en plus, on demande aux électeurs de parcourir des dizaines de kilomètres pour voter à l'urne ? On ne peut pas non plus compter sur le seul vote électronique, qui se heurte, en certains endroits, à la fracture numérique et à une incertitude quant à l'organisation optimale du vote par la société retenue. Dans le contexte actuel, cela va de soi, le renforcement de l'efficience du dispositif de vote électronique doit être garanti sur tous les continents.

Les conséquences ne sont pas nulles ; la charge de la masse salariale basculera sur les établissements, qui sont déjà en grande difficulté, puisque les postes de résidents ou de détachés sont transformés en des postes de recrutés locaux. La crise sanitaire frappe également de plein fouet le réseau de nos alliances françaises. Les 2 millions d'euros déployés ont certainement évité des fermetures, mais nous proposons une aide complémentaire, parce que la situation demeure critique.

ce réseau. Quant aux instituts français, dont le budget est stable par rapport à la loi de finances pour 2020, nous pensons qu'un fonds d'urgence les aiderait à traverser la crise. Ils ont puisé dans leur fonds de roulement, mais leur situation demeure extrêmement fragile. Nous avons l'immense honneur de posséder le premier réseau culturel au monde ; protégeons-le, chérissons-le Pour conclure, je veux rendre hommage à la mobilisation de l'ensemble du personnel- titulaires, contractuels ou recrutés locaux -de votre ministère, en poste à l'étranger comme en France, à commencer par vous, monsieur le ministre, sans oublier nos conseillers des Français de l'étranger et les associations, qui n'ont pourtant pas été épargnés. Cette mobilisation de nos réseaux et de nos relais locaux a permis le retour de plus de 370 000 Français. Elle assure la sécurité tant de nos ressortissants que de nos représentations. Elle fait vivre la citoyenneté de nos compatriotes, grâce au service public de nos consulats et aux élections qu'elle permet fait partager nos valeurs et notre langue dans notre réseau culturel et éducatif. Elle aide au développement des pays où nous sommes présents. L'une des leçons à tirer de la crise sanitaire qui nous touche est l'utilité d'un service public solide, qui protège et apporte son soutien quand tout semble s'écrouler. On ne peut pas compter sur le seul engagement et sur le seul dévouement du personnel, même si ce dernier a démontré qu'il avait su se mobiliser au pic de la crise et révéler ainsi la résilience de nos réseaux diplomatique, consulaire, culturel et éducatif.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le moins que l'on puisse dire, c'est que, depuis l'examen du dernier PLF, le contexte international ne s'est guère amélioré. Si l'élection de Joe Biden apporte un apaisement bienvenu à la relation transatlantique, elle n'entraînera sûrement pas le retour aux équilibres antérieurs, détruits par la pandémie mondiale qui a bouleversé notre planète. Les États puissances poussent leurs ambitions nationales dans de nombreux points du globe ; l'exemple des tensions stratégiques causées en Méditerranée orientale par les agissements de la Turquie, dont nous avons longuement débattu ces derniers jours, en est la preuve. Dans ce monde aux tensions exacerbées, le multilatéralisme, censé réguler la violence des relations internationales depuis la Seconde Guerre mondiale,

aiguise les appétits de pays qui entendent obtenir un « retour sur contributions ». C'est toutefois oublier la contribution de notre pays à la sécurité internationale,

Face à ce chaos géostratégique, la modestie des crédits du Quai d'Orsay nous apparaît dans sa cruelle réalité, même si le ministre multiplie, sur tous les fronts, les efforts pour faire entendre la voix de la France dans le monde. Bien sûr, l'augmentation de plus de 2 % des crédits de la mission que nous examinons aujourd'hui va dans le bon sens. Nous nous félicitons, monsieur le ministre, d'avoir été entendus sur plusieurs points, je voulais vous en faire part ; plusieurs évolutions que nous appelions de nos voeux Je pense en premier lieu à l'arrêt de la réforme Action publique 2022, qui prévoyait une importante réduction du personnel dans le cadre de la mutualisation des effectifs à l'étranger. réalisée à 80 %, est enfin interrompue, car vous avez bien voulu tirer les leçons de la pandémie ; les agents de votre ministère, éprouvés par cette réforme, ont été ont été essentiels pour le rapatriement des 370 000 Français coincés à l'étranger lors de la première vague de la covid. Je souhaite, moi aussi, leur rendre un hommage appuyé,

Les postes de présence diplomatique, au nombre de vingt-cinq, ont montré leurs limites. Ils ne sont fonctionnels qu'avec l'appui des réseaux régionaux, qui ne peuvent se déployer réellement que lorsque les transports aériens fonctionnent ; or ceux-ci sont interrompus, et cette réduction de format ne peut être étendue sans remettre en cause l'universalité de notre réseau. Nous recommandions également la « sincérisation » des crédits de cette mission, par la mise en place de mécanismes de couverture du risque de change et d'inflation,

nous les encourageons. Le doublement du nombre d'élèves dans les écoles et lycées français à l'étranger, annoncé en 2017 par le Président de la République, nécessite des moyens qui ne sont toujours pas au rendez-vous, malgré vos engagements, monsieur le ministre. C'est pourtant un volet essentiel de la politique de développement de la francophonie, à laquelle nous sommes tous attachés. Notre réseau éducatif à l'étranger a été fragilisé par la pandémie ; des mesures fortes sont donc attendues.

La rebudgétisation des crédits de sécurisation et d'entretien va dans le bon sens, mais le niveau est encore insuffisant au regard des besoins et des recommandations de notre commission. Il manque entre 20 millions et 40 millions d'euros pour l'entretien lourd des bâtiments. Les dépenses de sécurisation sont également loin d'avoir retrouvé le niveau préalable à leur basculement sur le compte d'affectation spéciale et à la mise en place d'un système de Gribouille : on vend

dans les moments difficiles de crises multiples que nous traversons et que vous gérez, votre engagement personnel est la garantie pour nous tous que les intérêts supérieurs de la France seront défendus. Nous voterons donc ce budget.

la crise pandémique a fortement affecté la vie de la communauté française à l'étranger. Permettez-moi de rendre hommage aux conseillers des Français de l'étranger, ainsi qu'au personnel des postes diplomatiques ou consulaires, qui viennent en aide à nos compatriotes en difficulté avec un grand dévouement, qui ont été particulièrement sollicités et qui ont répondu au-delà de toute attente. Alors que la crise perdure, il faut être vigilant à l'égard de nos compatriotes expatriés les plus fragiles. Un secours occasionnel de solidarité leur a été attribué par le plan de soutien.

leurs assurances, bref, le quotidien. Les critères d'attribution, totalement opaques et ne tenant pas compte des situations individuelles, sont évidemment la cause d'une si faible consommation des crédits. Le reliquat devrait être ajouté au budget de 2021 et les critères

La dotation de 410 000 euros qui leur est dédiée reste stable par rapport à 2020, alors que ces organismes ont été fortement sollicités pour venir en aide à nos compatriotes fragilisés par la crise sanitaire. Ce montant aurait dû être réévalué. Le réseau scolaire à l'étranger a été fortement affecté par la crise, mais il s'est montré résilient. On compte actuellement 531 établissements dans le réseau, soit 13 de plus que l'an passé.

Le budget de l'AEFE s'élèvera à 1 milliard d'euros, dont 417,1 millions d'euros de subvention ; il augmente de 9 millions d'euros pour financer la sécurisation des emprises immobilières. D'autre part, il a été constaté que l'on continue de transformer les postes de résidents en contrats de droit local, pour de simples raisons d'économies budgétaires, sans suffisamment tenir compte de l'expertise des enseignants ; c'est regrettable.

Sur les 50 millions d'euros de crédits du plan de soutien en faveur des établissements, environ la moitié a été consommée, l'essentiel étant consacré aux établissements du Liban, terriblement affectés par l'explosion intervenue à Beyrouth. Là encore se pose la question du report des crédits non consommés au budget de 2021. Le Président de la République a lancé un plan de développement de l'enseignement français à l'étranger. donner suite, l'AEFE a notamment besoin de retrouver sa capacité d'emprunt, afin de financer les projets immobiliers des établissements en gestion directe, au-delà des douze mois actuellement autorisés.

ans d'existence, après 169 prêts garantis, le dispositif de l'Anefe n'a jamais rien coûté l'État, ni en garantie ni en fonctionnement. Jamais l'État n'a été appelé en garantie ! De plus, le régime de l'Anefe présentait l'avantage de la rapidité d'instruction et de décision sur les dossiers.

quelque 577 alliances françaises, soit plus des deux tiers d'entre elles, étaient encore fermées au public ou en cessation d'activité et risquent de ne pas rouvrir si aucune aide ne leur est apportée. C'est une perte considérable pour la diffusion de la langue française et le rayonnement de la France. J'en viens maintenant à un sujet de préoccupation essentiel : les entreprises françaises créées localement par nos compatriotes expatriés, essentiellement des PME ou TPE, ont été les grandes oubliées du plan de relance. Aucune aide ne leur a été accordée, alors que leur contribution au développement de notre commerce extérieur et au rayonnement de la France est indéniable. Serge Babary, le président de la délégation sénatoriale aux entreprises, m'a confié

À la suite de l'attentat odieux contre Samuel Paty et des propos tenus sur la légalité des caricatures de Mahomet, des manifestations ont eu lieu contre le Président de la République et notre pays, et le boycott des produits français a été encouragé.

Monsieur le président, Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous, je suis totalement convaincu que la France a besoin d'une diplomatie forte. France a besoin d'une diplomatie forte pour faire face à la crise pandémique dans laquelle notre pays et notre continent se trouvent plongés depuis plusieurs

La France a besoin d'une diplomatie forte pour renforcer la souveraineté européenne, essentielle à la sienne propre, et pour mieux affirmer, sur la scène internationale, aux côtés de nos partenaires, un multilatéralisme nouveau,

Il va sans dire que la détermination des femmes et des hommes du Quai d'Orsay à assurer le retour de plusieurs centaines de milliers de Français- 370 000 exactement

des moyens humains, que je souhaite également pouvoir constater l'année prochaine, grâce à votre soutien, s'accompagne d'un renforcement de nos moyens de fonctionnement, en particulier sur trois sujets cruciaux, que j'ai eu l'occasion d'aborder avec vous à plusieurs reprises, notamment en commission, et que vous avez vous-mêmes évoqués tout à l'heure : l'immobilier, la sécurité et le numérique. Premièrement, nous avons changé de logiciel

le plan quadriennal de sécurisation de nos ambassades et des lycées français, dont la mise en oeuvre avait pris un peu de retard en raison de l'impact de la crise de la covid, sera achevé en 2021 pour les ambassades et en 2022 pour les lycées. Mais d'importants progrès ont déjà été accomplis, en pays en crise ont déjà été renforcées et sécurisées. Nous allons aussi permettre à l'AEFE d'assurer le renforcement de sa sécurité par un rebasage de 9 millions d'euros de sa subvention,

site étant exposé aux attaques en raison de la nature même du réseau informatique ; un besoin technique, car il est urgent de renforcer nos outils de mobilité et de communication ; enfin, un besoin de modernisation du service que nous rendons à nos usagers.

pour signifier notre soutien au multilatéralisme dans le domaine de la sécurité internationale. Nous avons ainsi financé davantage l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques,

cette stabilité masque l'effort financier important qui a été engagé en 2020 pour répondre aux conséquences économiques et sociales de la crise de la covid-19 pour les Français de l'étranger. Je rappelle que 200 millions

d'une aide exceptionnelle de subventions supplémentaires pour aider les familles à faire le choix de l'enseignement français à l'étranger, enfin, de 50 millions additionnels sur le programme 823, sous la forme d'avances de France Trésor, pour aider nos établissements. Je veux, à cet égard,

J'espère que nous pourrons aboutir à ce résultat. Cependant, les moyens de l'aide sociale seront, à budget constant, renforcés de 17 % en 2021 par rapport

la modernisation de notre action consulaire, grâce à une dématérialisation accrue des démarches administratives. Mme Conway-Mouret a appelé mon attention sur le vote par internet : celui-ci se concrétisera effectivement en 2021.

qui sera le centre de réponses téléphonique et courriel unique et dont l'expérimentation, initialement prévue en 2020, a dû être reportée d'un an. C'est aussi en 2021 que le registre de l'état civil électronique se mettra en place et que le développement

et l'impulsion d'une nouvelle dynamique de développement de l'enseignement français à l'étranger ; le rayonnement culturel et artistique, notamment par le renforcement de la diffusion et de l'exportation de nos industries culturelles et créatives

sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les points majeurs du PLF que je voulais évoquer auprès de vous. Voilà comment nous comptons employer ces moyens renforcés pour apporter des réponses diplomatiques, avec l'ensemble de nos partenaires, à toutes les grandes questions internationales qui engagent aujourd'hui le quotidien des Français, mais aussi l'avenir de notre pays. Je vous remercie de votre soutien. Nous allons

relais. Avant de retirer mon amendement au profit de celui de la commission, je veux dire que je ne suis absolument pas hostile au principe des ambassadeurs thématiques. Je crois même que, dans certains cas, ils peuvent être extrêmement utiles.

n'a fait qu'exacerber une situation déjà difficile. On touche aujourd'hui aux limites du financement des établissements du réseau de l'AEFE par les familles, car, lorsque ces dernières ne veulent

liés au protocole sanitaire et au déploiement du distanciel, inquiète les établissements. Le Gouvernement a profité des différentes lois de financement rectificatives de ce printemps pour abonder le réseau de d'un budget exceptionnel de 50 millions d'euros. En parallèle, le Trésor a été autorisé à faire une avance de 50 autres millions d'euros, mais il faut se souvenir d'où nous partons. Finalement, les familles participent aux alentours de 1,5 milliard d'euros au financement du réseau, estimé à environ 2 milliards d'euros. Aussi, on comprend mieux comment les frais d'inscription des établissements ont pu bondir de 25 % depuis 2012, pour atteindre 5 300 euros en moyenne. Nous sommes dans une situation d'urgence, que les 50 millions d'euros d'aides exceptionnelles et les 50 millions d'euros d'avances du Trésor ne pourront pas suffire à compenser. Notre amendement, s'il est forcément circonscrit financièrement, vise à faciliter l'instauration des protocoles sanitaires. C'est d'autant plus important que nous parlons d'un réseau dans 130 pays, qui doit donc s'adapter à 130 législations nationales et situations sanitaires. Or nous savons aussi que nous sommes dans une crise de long terme, avec des vagues épidémiques épidémiques successives touchant les différents pays. Cette complexité est encore aggravée par la multiplication des modes de gestion des établissements et des personnels, qui implique une influence différenciée du réseau de l'AEFE. Dans ces conditions, il nous semble essentiel de renforcer les crédits de ce réseau.

mettra fin à ces pratiques et, surtout, soutiendra les familles qui investissent et s'investissent très largement dans nos établissements. Cela dit,

combien l'engagement de la France dans l'OTAN est important et combien il assure notre propre liberté de parole. Vous avez pu vous en rendre compte ! L'adoption de

indispensables et de l'accompagnement puisse être pris en compte et que les familles se voient attribuer des volumes horaires et des quotités horaires correspondant à la réalité des besoins et des coûts. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ces crédits seraient prélevés sur l'action n° 01, Coordination de l'action diplomatique, du programme 105, « Action de la France dans le monde », et versés à l'action n° 02, Accès des élèves français au réseau de l'AEFE, du programme 151, « Français à l'étranger et affaires consulaires ». Quel est l'avis de la commission

visant à créer un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles- tremblements de terre, tsunamis ... -, de catastrophes sanitaires ou d'événements politiques majeurs- putsch, coups d'État

Monsieur le ministre,

Les instituts français et les alliances françaises sont un atout important en termes de coopération culturelle, de promotion du français et de diplomatie d'influence, nous le savons tous. Or l'épidémie de la covid-19 de la covid-19 et ses conséquences économiques ont considérablement fragilisé financièrement de nombreux instituts français et alliances. Certaines structures, qui ont connu des pertes financières considérables, pourraient ne pas rouvrir leurs portes. Nous sommes tous conscients du fait que l'apprentissage et la promotion de la langue française et du plurilinguisme constituent une nécessité et un atout dans la mondialisation, de même qu'un facteur de diversité indispensable.

pour continuer de développer le numérique et ainsi demeurer de véritables acteurs de la modernisation de la coopération culturelle et linguistique.

Ces 4 millions d'euros pourraient abonder les 9 millions d'euros de crédits affectés à la sécurisation des établissements et qui seront notoirement insuffisants. Cette hausse est indispensable pour éviter de recourir à une augmentation des frais de scolarité, déjà très élevés pour de nombreuses familles,

Cette hausse est également justifiée par l'objectif ambitieux affiché par le Président de la République de doubler d'ici à 2030 le nombre d'élèves scolarisés en français à l'étranger.

il convient dès à présent de préparer l'avenir et de tout faire pour que les étudiants étrangers choisissent notre pays et nos universités dynamiques pour accomplir leur cursus universitaire. Or, dans un monde où la compétition pour attirer les étudiants étrangers est forte, et compte tenu de l'augmentation des frais universitaires pour les étrangers, nous devons donner davantage de moyens à Campus France pour faire face à la concurrence internationale. chers collègues, je vous invite à voter cet amendement qui vise à abonder l'action n° 04, Enseignement supérieur et recherche, du programme 185, « Diplomatie culturelle et d'influence », à hauteur de 3 millions d'euros de crédits supplémentaires. Quel est l'avis de la commission

Même avis, monsieur le président. le Fonds citoyen commun créé par l'article 12 du traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle du 22 janvier 2019. Ce fonds est destiné à appuyer les projets conjoints d'acteurs de la société civile, notamment les initiatives citoyennes et les jumelages de communes.

C'est en effet au quotidien et par les actions promues par les citoyens ou par les communes au plus près des territoires que s'épanouira, à l'avenir, l'amitié entre nos deux pays, qui est plus essentielle encore que d'habitude dans les moments de crise que nous connaissons actuellement. Si ce fonds est primordial, son financement n'est pas à la hauteur. Mes chers collègues, je vous invite donc à le soutenir en le finançant à hauteur de 1 million d'euros.

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Action extérieure de l'État », figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix ces crédits, modifiés. J'appelle